Cette candidature sera ratifiée si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévu par notre règlement. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi relative à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs,

En effet, un service public, comme vous l'avez dit, madame la ministre, n'a pas vocation à être rentable : il doit répondre à un besoin et être financé à la hauteur de ce besoin. La mission d'intérêt général du transport ferroviaire est d'assurer un maillage suffisant du territoire national et de proposer un mode de transport non émetteur de gaz à effet de serre. Or, pour nous assurer de cela, nous devons dégager des ressources à même de désendetter la SNCF, de financer des investissements de rénovation ainsi que de nouveaux projets. Pour ce faire, en vertu du principe « pollueur-payeur », nous proposons que la route finance le rail. Ainsi, nous préconisons la renationalisation des autoroutes. La manne financière que constitue cette véritable rente s'élève à près de 2 milliards d'euros et serait beaucoup plus utile dans les caisses de SNCF Réseau que dans les poches des actionnaires d'Eiffage ou de Vinci. Dans la même logique, nous proposons la mise en oeuvre d'une écotaxe poids lourds, qui sera à même de lever 1 milliard d'euros supplémentaire et qui aura également un effet incitatif pour favoriser le fret ferroviaire. À travers cet amendement, nous proposons donc de pérenniser les financements du système ferroviaire, tout en renforçant l'effort de transition écologique dans le secteur du transport. Quel

Le Gouvernement a déjà conduit un certain nombre de réflexions dans le cadre des Assises nationales de la mobilité et à travers les rapports de MM. Duron et Spinetta. Nous espérons que la loi d'orientation sur les mobilités proposera des solutions concrètes dans ce domaine.

du Gouvernement ? Je vous confirme que je suis engagée dans une réforme globale du secteur des transports qui vise tout à la fois à retrouver une trajectoire économique équilibrée pour notre système ferroviaire et à assurer un financement pérenne de nos infrastructures à la hauteur des besoins, dans une démarche sincère. La future loi de programmation qui sera débattue prochainement sera équilibrée en ressources et en dépenses. Dans le cadre notamment des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, des propositions ont été formulées sur le financement de notre politique de transport. Nous n'en sommes donc plus à la remise de rapports, mais à traduire

Nous voulons ainsi interdire le recours aux contrats de partenariat public-privé pour le financement, la construction ou la transformation, l'entretien, la maintenance, l'exploitation ou la gestion d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels nécessaires pour les infrastructures de transport terrestre. Il s'agit ainsi de réaffirmer la nécessaire maîtrise publique des infrastructures de transport et de tirer toutes les conséquences de l'expérience du recours au partenariat public-privé, souvent plus coûteux pour la collectivité et les usagers et moins performant en termes de services. Dans le cadre d'une volonté affirmée de mieux maîtriser les dépenses engagées en faveur du réseau ferroviaire, il convient de tirer les conséquences de ces expériences coûteuses pour les deniers publics. Il y a une semaine, le 20 mars dernier, la Cour des comptes européenne a présenté un rapport mettant en doute les avantages de ces opérations. Elle relève Elle relève que les PPP « ne peuvent être considérés comme une option économiquement viable pour la fourniture d'infrastructures publiques », à cause « du manque de clarté des politiques et des stratégies, d'analyses inappropriées, de la comptabilisation des PPP hors bilan et d'une répartition déséquilibrée des risques ». son rapport que la majorité des PPP se sont montrés inefficaces : sept des neuf projets achevés ont accusé des retards allant jusqu'à cinquante-deux mois et ont connu une forte augmentation des coûts. précise également : « Des fonds publics supplémentaires d'un montant de près de 1,5 milliard d'euros ont été nécessaires à l'achèvement des cinq autoroutes auditées en Grèce et en Espagne. L'UE a fourni quelque 30 % de ce montant. » Le rapport conclut en indiquant que « ces dépenses ont été inefficaces dans la mesure où les avantages économiques potentiels n'ont pas été obtenus ». Toutes les analyses sont donc aujourd'hui concordantes pour nous alerter sur ce type de montage. Cet amendement en tire les conséquences. Quel est l'avis de la commission ? Cet

Il s'agit d'un élément important de nos propositions pour de nouveaux financements en faveur de notre système ferroviaire, nouveaux financements que nous considérons comme particulièrement urgents. Nous estimons en effet que toute réforme ferroviaire devrait avoir pour objectif prioritaire de donner les moyens aux acteurs ferroviaires de remplir leurs missions d'intérêt général. Je rappelle, dans ce cadre, que les régions sont actuellement les seules autorités organisatrices qui ne perçoivent pas de versement transport. Les collectivités territoriales situées en périmètre urbain en bénéficient, tout comme la région d'Île-de-France, qui dispose d'un régime spécifique. Il faut, nous semble-t-il, mettre fin à cette injustice. Il paraît également opportun que l'ensemble des entreprises qui bénéficient, pour leurs salariés et leurs clients, de bonnes conditions de mobilité s'engagent à participer à ce financement. Avec la mise en place d'un versement transport régional, les régions bénéficieraient d'une ressource propre, pérenne et dynamique, permettant d'engager le nécessaire renouvellement du matériel ferroviaire et d'améliorer l'offre de transport collectif. Il ne s'agit pas d'une bagatelle, puisque le produit attendu pourrait atteindre 700 millions d'euros, autant d'argent utile pour le développement du transport régional, plus utile, nous semble-t-il, qu'une ouverture à la concurrence. Ces ressources sont nécessaires, alors que les régions seraient appelées à récupérer le matériel roulant et les ateliers de maintenance, selon cette proposition de loi. Concrètement, le versement transport régional que nous proposons pourra être porté à un taux régional plafonné à 0,3 % des salaires sur les zones situées en dehors du ressort territorial de l'autorité organisatrice de mobilité- c'est ce qu'on appelait auparavant le périmètre de transports urbains -, avec un taux additionnel, dans le ressort territorial de cette autorité, plafonné, lui, à 0,2 %. Cette question est sur la table depuis de nombreuses années. Il faut la trancher et accompagner les régions dans leurs compétences. Quel ? Cet amendement vise à généraliser le versement transport dans les zones qui ne sont pas couvertes par une autorité organisatrice de mobilité et à créer un versement transport additionnel au profit des régions, afin de leur permettre de financer le développement du transport ferroviaire de voyageurs. Examiner un tel amendement dans le cadre de cette proposition de loi est à mon sens prématuré, puisque les questions relatives à la couverture de l'ensemble du territoire par une autorité organisatrice de transport et à la généralisation du versement transport seront traitées dans le cadre du projet de loi d'orientation sur les mobilités,

Mme Éliane Assassi. Cet amendement tend à appliquer aux transports publics urbains et interurbains de voyageurs, notamment aux transports publics soumis à des obligations de service public comme les TER et les TET, le taux dévolu aux produits de première nécessité, soit 5,5 %, en considération de leur rôle social essentiel et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique. Un tel taux allégerait également la facture pour les régions et les intercommunalités. Nous reprenons ici l'article 3 de notre proposition de loi

du Sénat. De plus, il correspond à une sollicitation de l'Association des régions de France. L'adoption de cet amendement permettrait d'envoyer un signal clair en faveur du développement des transports régionaux.

reprise de la dette, qui obère toute possibilité d'investissement dans les réseaux et donc le développement d'une nouvelle offre de transport ; financements nouveaux pour les régions, qui assurent les transports du quotidien ; suppression des partenariats public-privé, qui sont un gouffre pour les deniers publics développement du fret ferroviaire comme une alternative au transport par camion afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais, cela, ni la majorité sénatoriale ni le Gouvernement ne le souhaitent, et tous ces amendements ont été rejetés d'un revers de main. On en parlera plus tard, avez-vous dit Vous n'avez qu'un mot à la bouche : concurrence. Comme s'il s'agissait d'une formule magique ! Mais en quoi le changement d'opérateurs sera-t-il bénéfique aux usagers si les réseaux continuent de se dégrader, entraînant, quel que soit l'opérateur, ralentissements et autres désagréments ? En quoi l'ouverture à la concurrence et, donc, la perte du monopole de la SNCF sont-elles des réponses aux besoins nouveaux de mobilité, puisqu'il y a fort à craindre que les nouvelles compagnies, comme c'est absolument normal, ne se focalisent sur les axes rentables laissant le soin aux autres d'assumer des axes tout aussi structurants, mais moins usités Quel progrès pour la sécurité ? Quel progrès pour la tarification ? Cela va conduire la SNCF elle-même à abandonner certaines des dessertes, vu qu'elle ne sera plus liée, par son monopole, à une obligation de faire, comme le code de transports l'indique, selon « les principes du service public En réalité, cela fait longtemps que les gouvernements successifs préparent cette réforme. On a affaibli la SNCF en la coupant en tronçons, on l'a fragilisée en empêchant la péréquation entre les différentes activités, en organisant l'assèchement des ressources, pour pouvoir maintenant l'accuser de tous les dysfonctionnements, alors même que c'est l'État qui a organisé sa faillite. Aujourd'hui, on franchit un pas supplémentaire dans l'affaiblissement de l'entreprise historique avec l'ouverture à la concurrence, qui prépare sa privatisation et la fin du service public ferroviaire.

Je rappelle que l'ouverture à la concurrence a été décidée sous le précédent quinquennat. Elle est attendue par les régions pour offrir un meilleur service aux voyageurs.

alinéa de l'article L. 2141-1 du code des transports en matière de gestion des gares de voyageurs. Il ne paraît donc pas inopportun de l'imposer également à la mission d'exploitation des services de transport ferroviaire. Quel est l'avis de la commission ? commission ? Cet amendement vise à préciser que SNCF Mobilités exploite des services de transport ferroviaire de façon transparente, comme il est aujourd'hui indiqué pour les gares que SNCF Mobilités les exploite de façon transparente et non discriminatoire ». Cette mention se justifie, pour les gares, par la nécessité de favoriser l'accès de toutes les entreprises à ces installations, alors que Gares & Connexions est encore une direction de SNCF Mobilités. Je suis plus réservé sur la reprise partielle de cette expression pour l'exploitation, par SNCF Mobilités, de services de transport qui pourront être, demain, librement organisés. L'opérateur sera alors dans la même situation que les autres entreprises ferroviaires, et la portée de cette précision est difficile à apprécier. Je suis en revanche tout à fait d'accord sur le fait que SNCF Mobilités doit être transparente vis-à-vis des autorités organisatrices. Sur ce dernier point, je considère que l'amendement est satisfait par le dispositif contraignant d'obligation de transmission d'informations prévu à l'article 7. En conséquence,

Gares & Connexions. Cette branche de SNCF Mobilités, créée en 2009, a vu régulièrement son autonomie renforcée. Les économistes qualifient de facilités essentielles ce genre de fonctions, dans la mesure où elles sont difficilement reproductibles. Pourtant, elles sont indispensables aux opérateurs pour exercer leurs activités. Elles peuvent être vues comme un monopole naturel et exiger, pour cette raison même, des caractéristiques bien particulières, par exemple en matière de propriété du capital- j'y reviendrai. Le rattachement de Gares & Connexions à SNCF Mobilités est très critiqué par ceux qui pensent que ce rattachement

évoquait différents scénarios, dont le transfert à SNCF Réseau, avec la création d'un établissement public indépendant. Les auteurs de la proposition de loi envisagent de transformer Gares & Connexions en SA rattachée à l'EPIC de tête SNCF. Une telle proposition est loin de faire l'unanimité ; nous n'y sommes pas non plus favorables. Quel est l'avis de la commission ? Il y de la commission ? Il y a consensus sur la nécessité de séparer la gestion des gares de SNCF Mobilités dans le contexte de l'ouverture à la concurrence.

éminents collègues que la commission peut, le cas échéant, demander que l'on réexamine un amendement de coordination si l'amendement principal est adopté. En cela, M. Cornu a tout à fait raison. Il se trouve que le déroulement de la séance fait que l'on voit l'accessoire avant le principal,

M. Guillaume Gontard. Cet article prévoit que les services conventionnés ferroviaires peuvent être assurés par la voie d'un marché public ou d'un contrat de concession par une entreprise autre que l'entreprise publique SNCF Mobilités. Nous ne partageons pas cette volonté d'aller vers l'ouverture à la concurrence des transports dits « conventionnés », c'est-à-dire principalement les services régionaux et les trains d'équilibre du territoire. En effet, il s'agit non seulement de l'offre la plus structurante pour les territoires, mais aussi de l'offre la moins rentable économiquement parlant. Il n'est donc pas sûr que l'exploitation de ces lignes par des entreprises privées, guidées par la volonté du profit plus que par toute autre considération, soit une bonne nouvelle pour les usagers. Au total, ces derniers risquent surtout de voir les dessertes les moins rentables abandonnées et le prix des billets augmenter. Tel a été le cas pour tous les services publics libéralisés : l'énergie, les télécommunications, et j'en passe. et j'en passe. Les TET ainsi que les TER sont des facteurs de cohésion et de désenclavement territorial. Ils relèvent donc de l'intérêt général. Nous l'avons dit, nous craignons que cette ouverture à la concurrence ne soit l'occasion, une nouvelle fois, d'abandonner un certain nombre de lignes et de dessertes. l'État fait pression sur les régions pour la reprise des lignes du quotidien, puisqu'il leur demande de recenser les besoins et donc, en creux, de définir les axes inutiles. Il aurait été plus opportun, comme nous l'avons proposé par nos amendements, de prévoir de nouvelles ressources pour développer ces offres de transport. également plus opportun de conserver un opérateur public en situation de monopole, permettant d'organiser la péréquation sur l'ensemble du territoire national et exerçant cette mission de service public.

Nous considérons, à l'inverse, qu'il aurait fallu se fonder sur les exceptions prévues par le règlement OSP, sur la nature même de ce réseau dont l'exploitation revêt une dimension d'intérêt général en permettant l'aménagement du territoire et en offrant une solution de substitution à la voiture. Pour l'ensemble de ces

plus, je ne peux pas laisser dire que les régions ou l'État voudraient, à cette occasion, réduire le service public. Les régions ont la responsabilité d'organiser les TER. Si elles demandent l'ouverture à la concurrence, c'est pour offrir

si les trains n'arrivent plus à l'heure, si certaines lignes n'ont pas été entretenues et si la SNCF s'est transformée, au fil du temps, en tonneau des Danaïdes

Avis défavorable. La loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs s'appliquera aux nouveaux entrants sans qu'il soit nécessaire d'y faire référence dans le code des transports.

en réalité, le service minimum n'est pas mis en oeuvre. Je ne vois pas les pouvoirs publics en arriver à la réquisition pour le faire appliquer. Il faut donc trouver d'autres modalités. La loi de 2007 était une étape.

couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale. Même si ce dispositif est encadré, nous nous interrogeons sur cette disposition, qui est très contraignante à l'égard de l'opérateur public. Certaines données peuvent relever du secret des

M. Jean-Pierre Corbisez. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs doit être anticipée et ses modalités doivent être préparées dans les moindres détails, à la fois pour ne pas pénaliser inutilement l'opérateur historique en transmettant des données sensibles,

L'article 2 encadre la transmission aux candidats, par les autorités organisatrices de transport, des informations nécessaires à l'appel d'offres. Le règlement OSP prévoit que « les autorités compétentes mettent à la disposition de toutes les parties intéressées des informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, tout en garantissant la protection légitime des informations commerciales confidentielles ». La présente proposition de loi reprend d'ailleurs ces termes. Il s'agit donc, par cet amendement, de renforcer la protection du secret industriel et commercial de notre entreprise historique en précisant que seules sont transmises les données strictement nécessaires pour éviter les distorsions de concurrence. Quel

entre, d'une part, la protection légitime du secret industriel et commercial et, d'autre part, la nécessité de permettre à l'ensemble des candidats d'avoir les informations indispensables à la présentation d'une offre. À défaut, SNCF Mobilités possèdera toujours un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants et ceux-ci ne pourront pas présenter de plan de transport sérieux. C'est la raison pour laquelle l'article 2 de la proposition de loi prévoit la transmission de données couvertes par le secret industriel et commercial, mais de façon proportionnée et encadrée. Cette transmission n'aura lieu que si cela est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence. Elle aura lieu dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'État pris après avis de l'ARAFER, pour protéger la confidentialité de ces données. Certaines informations devront par exemple être présentées par fourchette de valeurs, ou ne pourront être consultées que dans une salle spécifique,, etc. Ce procédé n'a rien d'incongru ni d'exceptionnel. L'ordonnance relative aux contrats de concession prévoit ainsi que « l'autorité concédante peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées et que « les autorités concédantes peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'elles communiquent dans le cadre de la procédure de passation du contrat de concession

Ces deux amendements visent à préciser les informations qui doivent être transmises en amont de la préparation des appels d'offres. Il s'agit bel et bien d'un sujet sensible : il faut trouver un bon équilibre entre l'information de l'autorité organisatrice, l'équité de la concurrence et la protection des savoir-faire des entreprises ferroviaires, en particulier de la SNCF. Sur ces sujets, les concertations sont en cours. Dans l'attente de leurs résultats, je m'en remets à la sagesse du Sénat.

l'opérateur est tenu de les fournir selon un standard ouvert et aisément réutilisable. Cette ouverture des données publiques semble être un gage de bonne foi à l'égard des utilisateurs : chacun doit disposer de l'ensemble des informations publiques dans de bonnes conditions pour pouvoir se faire son opinion.

cet article en interdit l'utilisation. Cette interdiction est d'autant plus surprenante qu'il n'en est fait nullement mention dans l'exposé des motifs. c'est l'application du paragraphe 4 de l'article 5 de ce règlement : « Sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemins de fer : « Lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concernés, et notamment leur taille, les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau, son isolement technique et géographique et les services couverts par le contrat Lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent

Les dispositions du présent article excluant toute possibilité de préservation du service public et écartant ainsi l'application du règlement OSP nous semblent particulièrement dangereuses et dogmatiques. Nous en proposons donc la suppression, et nous appelons le Gouvernement à se saisir des finesses du règlement OSP

peuvent décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs » aux transports par chemins de fer, à l'exception d'autres modes ferroviaires, comme le métro ou le tramway. La durée de ces contrats ne pourra généralement pas dépasser dix ans. Ces dispositions peuvent s'appliquer du 3 décembre 2019 au 24 décembre 2023, soit pendant quatre ans. Elles permettent aux autorités compétentes, en l'occurrence les régions, de choisir la procédure d'attribution directe de contrats de service public ou la procédure de mise en concurrence. Ce choix possible d'une ouverture progressive à la concurrence, étalée entre 2019 et 2023, doit être préservé. Tel est le sens de notre amendement. Par ailleurs, le même article 5 du règlement OSP prévoit d'autres dérogations, plus spécifiques, à la procédure de mise en concurrence. Les paragraphes 3, 4, 4 et 4 , par exemple, traitent des situations structurelles et géographiques particulières des réseaux et du cas des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'attribution directe a pour effet d'améliorer la qualité des services, le rapport coût-efficacité ou les deux. Là aussi, pourquoi ne pas préserver ces dérogations, qui permettent de procéder par attribution directe à SNCF Mobilités sous certaines conditions, après 2023 ? Dans certains cas, cette solution pourrait être utile. Quoi qu'il en soit, ne privons pas les régions de cette possibilité de repousser, au-delà de 2023, l'ouverture à la concurrence et de s'adapter parfaitement. C'est justement le sens de la décentralisation., il nous semble utile de laisser le choix aux autorités organisatrices qui le souhaitent de continuer à attribuer directement à SNCF Mobilités un contrat de service public sans recourir à la procédure de mise en concurrence, et ce au-delà de 2023. Ainsi, en Île-de-France, vu l'état du réseau, le rapport Spinetta préconise de repousser très loin l'ouverture à

permettant aux autorités organisatrices qui le décident d'attribuer directement des contrats de service public entre 2019 et 2023. La durée de ces contrats ne pourra en aucun cas dépasser dix ans.

Les amendements n 14 rectifié et 47 visent à permettre aux autorités organisatrices de mettre en oeuvre l'ensemble des dérogations à l'obligation de mise en concurrence prévues par le règlement n° 1370/2007 et que les États membres sont libres de reprendre dans leur droit national ou non. Cette mesure est à l'opposé de la démarche volontariste qui est celle de cette proposition de loi. Il ne s'agit pas de verser dans la « surtransposition », mais de faire des choix clairs, en faveur de l'ouverture à la concurrence ou non. Je citerai, là encore, l'étude de l'ARAFER publiée mardi dernier ; elle indique que certaines des dérogations prévues par le règlement européen ont des conditions d'application très peu définies et pourraient ainsi être utilisées pour retarder, de fait, la mise en oeuvre de l'ouverture à la concurrence. Nous estimons que l'ouverture à la concurrence va améliorer la qualité du service rendu aux voyageurs et réduire les coûts. Nous souhaitons, en conséquence, qu'elle devienne la règle. J'ai néanmoins entendu les acteurs concernés et compris que certaines régions souhaitent profiter de la possibilité offerte par le règlement européen d'attendre 2023 pour ouvrir l'ensemble de leurs services à la concurrence.

du Gouvernement ? Il me semble que des modalités d'ouverture à la concurrence qui ne permettraient pas une attribution directe au-delà de décembre 2019

est de proposer la mise en place d'une ouverture progressive à la concurrence en tenant compte des demandes des régions. Dans l'attente des résultats de cette concertation, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur les trois amendements.

Le présent texte ne reprend donc aucune des dérogations autorisées par le quatrième paquet ferroviaire et permettant à une autorité organisatrice de transport de s'exonérer d'une procédure de mise en concurrence. » Le principe est, pour nous, l'ouverture à la concurrence.

passait ce thème totalement sous silence. En revanche, le rapport d'information qui avait été examiné par la commission des affaires européennes le 17 juillet 2013 comportait la proposition suivante : « Laisser à chaque État membre la faculté d'ouvrir un marché de délégation de service public incluant

que « les périmètres des marchés de délégation de service public doivent pouvoir inclure, dans une perspective d'aménagement du territoire, des liaisons déficitaires et des liaisons rentables de telle sorte que leur exploitation globale soit équilibrée au moment de la passation du marché ». Cette insistance argumentée fut couronnée de succès, puisque le règlement définitif adopté le 14 décembre 2016 par les instances communautaires autorise l'autorité compétente à spécifier des obligations de service public en regroupant

Il me semble toutefois utile d'apporter une clarification rédactionnelle afin de parfaire l'intelligibilité de la loi que nous sommes en train d'écrire. En effet, un lecteur quelque peu peu distrait pourrait croire que le champ des contrats de service public spécialement destinés à satisfaire les besoins d'aménagement du territoire devrait nécessairement inclure une liaison à grande vitesse. Je ne conteste nullement l'intérêt de contrats de service public associant au moins une ligne à grande vitesse et des liaisons ferroviaires locales à l'équilibre économique précaire, mais l'aménagement du territoire peut aussi conduire les autorités compétentes à conclure des contrats de service public associant des liaisons locales déficitaires à des lignes de transport ferroviaire équilibrant leurs comptes sans relever pour autant de la grande vitesse. Cette possibilité résulte du règlement adopté le 14 décembre 2016. Celui-ci étant d'application directe, l'amendement n° 44

Gontard. Le présent article prévoit la conclusion, par l'État, de contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes incluant des services à grande vitesse, pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire.

En effet, au travers de ces contrats de service public, il s'agit d'obliger les opérateurs à mixer services à grande vitesse rentables et services non rentables, pour permettre la continuité de la desserte, l'aménagement du territoire, mais aussi la péréquation entre les différentes offres. autant de missions qui étaient dévolues à SNCF Mobilités à une échelle plus pertinente, permettant une réelle péréquation. Pour notre part, même si nous comprenons les intentions des auteurs de la proposition de loi, nous estimons que ces garde-fous ne sont que des emplâtres sur une jambe de bois, d'autant que cette volonté de promouvoir l'aménagement du territoire ne concerne aucunement les transports régionaux, les petites lignes largement menacées par le rapport Spinetta, mais simplement les lignes à grande vitesse.

autant d'éléments qui nous confortent dans notre analyse que l'ouverture à la concurrence sera instrumentalisée afin d'abandonner un certain nombre de lignes jugées trop peu rentables. Il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, madame la ministre, de multiplier les offres : cette multiplication n'interviendra que sur les axes rentables ; ailleurs, ce sont des déserts ferroviaires que vous préparez. Il s'agit, une nouvelle fois, d'affaiblir la SNCF, selon un schéma où l'on privatise les profits et où l'on socialise les pertes. Nous nous inscrivons en faux contre cette conception. Le service public ferroviaire est un service en réseau qui doit permettre le maillage de l'ensemble du territoire, assuré par une offre cohérente et financé grâce à un soutien public et une péréquation tarifaire.

en cours. Il faudra aussi prendre en compte le cas des régions qui conventionnent un certain nombre de dessertes TGV

auteurs de l'amendement proposent que l'État présente à la Conférence nationale des territoires et aux commissions compétentes du Parlement sa stratégie pour la conclusion des contrats de service public. de service public. Je rappelle que la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire a créé un schéma national des transports, censé fixer les orientations de l'État

Ce dispositif vise à corriger la tendance naturelle du marché à l'écrémage : vous organisez une sorte de pour prendre en compte les exigences d'aménagement du territoire.

Seule une entreprise publique, chargée de missions de service public, peut satisfaire des exigences d'aménagement du territoire, en mettant en oeuvre un principe de péréquation nationale pour garantir en tout point du territoire un service public assurant l'effectivité du droit à la mobilité pour tous. Sans une telle implantation nationale, les entreprises n'auront pas les reins assez solides pour assumer l'exploitation de lignes fortement déficitaires. En outre, en l'absence d'étude d'impact,

ou ces dispositions et les limitations à la concurrence qu'elles induisent seront-elles utilisées avec parcimonie ? M. le rapporteur nous a donné des éléments de réponse en commission, puisque l'article 4 a été récrit afin d'expliciter que l'objectif n'est pas de couvrir l'ensemble du réseau.

rectifié vise à intégrer dans le champ de la proposition de loi les dispositions d'exception prévues au 8 de l'article 1 de la directive européenne 2016/2370. Il s'agit de ne pas surtransposer le texte européen, en autorisant le recours aux exceptions prévues par le règlement pour des pour des attributions dans certaines circonstances exceptionnelles : ligne isolée de moins de 500 kilomètres avec un écartement des voies différent de celui du réseau national, liaison avec un autre pays non régi par les règles de l'Union européenne ou gestion de l'infrastructure par un gestionnaire différent de celui du principal réseau.

Les dérogations qui pourraient être nécessaires en application du règlement sur les obligations de service public font actuellement l'objet de concertations avec, notamment, les

L'article 7 prévoit un dispositif contraignant pour permettre aux autorités organisatrices de transport d'obtenir de SNCF Mobilités et de SNCF Réseau des informations nécessaires à l'organisation des services ferroviaires. ferroviaires. Nous comprenons bien que, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et pour préparer leurs appels d'offres, les régions devront pouvoir disposer de certaines informations. Pour autant, l'article prévoit la transmission obligatoire de toute information jugée nécessaire par l'autorité organisatrice de transport, sans que puisse y faire obstacle le secret en matière industrielle et commerciale. En conséquence, l'autorité organisatrice de transport devra prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des tiers non autorisés n'aient accès à des données dont le caractère serait confidentiel.

lieu à la transmission d'informations sensibles à de nouveaux entrants. Comment faire pour ne pas affaiblir l'opérateur historique et préserver ses intérêts dans la compétition mondiale, si l'on livre des informations et des savoir-faire acquis de longue date, résultant parfois de nombreuses années d'ingénierie, de recherches technologiques ou de recherches sur les types d'organisation permettant d'optimiser l'ensemble des fonctionnements et des coûts l'heure où le Parlement s'apprête à renforcer le secret des affaires, les auteurs de l'amendement s'interrogent sur la nécessité d'obliger l'opérateur historique public SNCF Mobilités à fournir ce type particulier d'informations qui relèvent de la confidentialité et de la protection des intérêts L'ouverture à la concurrence ne doit pas permettre aux nouveaux entrants de récupérer sans aucune réciprocité des savoir-faire et des informations confidentiels leur conférant d'entrée de jeu un avantage concurrentiel sur l'opérateur historique. Dans de telles conditions, l'ouverture à la concurrence constitue un jeu de dupes

Les interrogations des auteurs de l'amendement au sujet de la protection de ce secret sont évidemment légitimes. Je rappellerai tout d'abord que le dispositif de transmission des informations prévu à l'article 7 est proportionné et encadré.

Il ne s'agit donc pas de livrer des savoir-faire aux nouveaux entrants. D'ailleurs, le périmètre des données que les autorités organisatrices de transport transmettront à leur tour aux candidats à un appel d'offres sera plus réduit et lui aussi très encadré, par l'article 2. si un agent de l'autorité organisatrice de transport divulgue ces données de façon indue, il s'expose à une sanction pénale lourde. L'accès des autorités organisatrices de transport à un certain nombre d'informations est essentiel pour qu'elles puissent exercer leurs missions correctement. Aujourd'hui déjà, elles ne parviennent pas à obtenir de la SNCF les informations dont elles ont besoin, alors même que les services ferroviaires ne sont pas ouverts à la concurrence. Le secret industriel et commercial est souvent invoqué par l'opérateur pour refuser la transmission des informations nécessaires, alors qu'il s'agit de services publics majoritairement financés par les régions. Ce besoin d'informations sera encore accru dans le contexte de l'ouverture à la concurrence, car les informations recueillies permettront aux autorités organisatrices de transport de définir leurs contrats de service public. C'est un point sur lequel l'ARAFER insiste particulièrement dans son étude sur les conditions d'une ouverture à la concurrence efficace des services conventionnés : « Il est organisatrices de transport disposent, par principe, d'un droit d'accès à toute information détenue par l'opérateur sortant relative à l'exécution du service conventionné. Pour ce faire, une disposition législative édictant le principe selon lequel l'autorité organisatrice de transport peut exiger de l'opérateur sortant qu'il fournisse toute information économique, financière ou technique relative à l'exécution du service qui lui est confié est indispensable, afin que le secret en matière industrielle et commerciale ne puisse faire obstacle à la transmission de ces données. » Compte tenu de tous ces éléments, j'émets un avis défavorable sur l'amendement n° 50.

Éliane Assassi, sur l'article. Cet article tire les conséquences de l'ouverture à la concurrence des services conventionnés en permettant le transfert des cheminots vers les entreprises qui auront remporté le marché.

des différents marchés, de plus en plus de cheminots statutaires se trouveront écartés de leur entreprise. Une telle démarche condamne évidemment le statut à petit feu. Pis, l'avis de ces cheminots comptera peu dans le processus, car s'ils refusent le transfert, il sera purement et simplement mis fin à leur contrat.

Toutes ces dispositions sont scandaleuses et prolongent au fond le plan social engagé à la SNCF, où le nombre d'emplois publics diminue constamment depuis des décennies. Les pouvoirs publics font des cheminots les boucs émissaires de tous les maux qui affectent le transport ferroviaire. C'est un chiffon rouge bien utile

Le peu de concertation avec les syndicats sur cette proposition de loi est éloquent : seuls deux des quatre syndicats représentatifs ont été ont été auditionnés par le rapporteur. Plus globalement, au lieu de tirer les conditions sociales vers le bas et d'organiser le social entre salariés du rail, ainsi qu'entre salariés du rail

la négociation avec les partenaires sociaux et à ouvrir la voie à une réforme ferroviaire qui ne signe pas la condamnation du service public et permette d'en finir avec l'avantage concurrentiel de la route. L'amendement n° 17, présenté par Mme Assassi,

objet indique que ses auteurs s'opposent à une attaque frontale contre le statut de cheminot. Or, dois-je le rappeler, la proposition de loi ne prévoit pas la fin du statut de cheminot. Elle fixe le cadre du transfert des salariés de SNCF Mobilités vers les opérateurs alternatifs qui remporteront des appels d'offres en vue d'exploiter des services ferroviaires. Pourquoi est-il nécessaire d'organiser le transfert des salariés en cas d'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire ? Tout simplement parce qu'il serait difficilement concevable que SNCF Mobilités, en perdant l'exploitation de certaines lignes, se retrouve avec des salariés en surnombre au regard de ses besoins,

compétents pour exploiter le service ferroviaire concerné permettra d'éviter que le nouvel entrant doive recruter et former des salariés à cette fin, ce qui prend beaucoup de temps. Cela garantira la fluidité du changement d'opérateur, au bénéfice des usagers. Au demeurant, je rappelle que le transfert de salariés en cas de perte de marché, qui est un principe s'appliquant dans de nombreux secteurs d'activité, dont celui des transports, est avant tout conçu pour protéger les salariés, en évitant que ceux-ci ne perdent leur emploi au sein de l'entreprise ayant perdu le contrat.

L'enjeu aujourd'hui est de préparer une ouverture à la concurrence progressive qui soit un succès pour les voyageurs,

Ne pas prendre en compte cette réalité et refuser d'aborder ces sujets ne rend pas service à la SNCF ni aux cheminots. Cela étant dit, dans l'attente du résultat des concertations en cours, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

par catégorie d'emploi, devant faire l'objet d'un transfert. Ce nombre est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l'appel d'offres. Deuxième étape, les Deuxième étape, les entreprises ferroviaires sortantes définissent à partir de ce périmètre la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d'affectation au service transféré, après consultation des représentants des salariés et avis de l'autorité organisatrice de transport. Troisième étape, les salariés ne figurant pas sur cette liste en raison d'un degré d'affectation moins important au service transféré peuvent se porter volontaires pour être transférés à l'entreprise ferroviaire entrante, et ainsi remplacer les salariés figurant sur la liste s'ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles que

Au terme de cette procédure, un salarié pourra être transféré sans son consentement. Pis, la possibilité que les contrats de cheminot puissent prendre fin de plein droit est ouverte en cas de refus du transfert. Une telle disposition méconnaît et bafoue les droits élémentaires attachés au statut de cheminot, qui ne prévoit la fin d'un contrat que pour démission, retraite, licenciement pour motif disciplinaire, licenciement pour inaptitude ou rupture conventionnelle. Une telle procédure ouvre la voie à un plan de licenciement massif chez l'opérateur historique, qui devrait être assujetti à une obligation de reclassement des salariés ne souhaitant pas être transférés. Elle fragilisera le statut des cheminots et ouvre la voie à une précarisation des salariés du rail.

notamment ceux d'entre eux qui, du fait de leur fonction ou de leur métier, seraient directement ou indirectement concernés par le transfert d'activité ? Ce droit d'option devrait pouvoir s'accompagner de la continuité de certains droits sociaux, autrement dit d'une continuité d'une continuité juridique dans l'appartenance au statut ou, pour le dire encore autrement et de manière plus imagée, de dispositions sociales incluses dans ce fameux « sac à dos social ». Concrètement, l'article prévoit que les salariés transférés seront en priorité désignés sur le fondement du volontariat. Si le nombre des salariés volontaires est inférieur au nombre de salariés à transférer,

prévoit une procédure en plusieurs étapes. Première étape, l'autorité organisatrice de transport définit le nombre de salariés devant faire l'objet d'un transfert. Celui-ci est communiqué aux entreprises souhaitant candidater à l'appel d'offres. à l'appel d'offres. Deuxième étape, les entreprises ferroviaires sortantes définissent à partir de ce périmètre la liste nominative des salariés à transférer en fonction de leur degré d'affectation au service transféré, après consultation des représentants des salariés et avis de l'autorité organisatrice de transport. Troisième étape, les salariés qui sont volontaires peuvent demander à remplacer les salariés devant faire l'objet d'un transfert obligatoire s'ils possèdent les mêmes qualifications professionnelles qu'eux. Enfin et surtout, les salariés devant faire l'objet d'un transfert peuvent faire valoir un droit d'option et refuser le transfert. En contrepartie, ils seront tenus d'accepter une mobilité géographique proposée par leur employeur, cette proposition devant leur être communiquée dans un délai raisonnable.

en contrepartie d'un refus du transfert est légitime, puisqu'il faut bien que les salariés dont le service ferroviaire a été transféré à une autre entreprise puissent être affectés

Dans ce cadre, sur le fondement de la liste des salariés transférables, les salariés concernés seraient proposés pour un transfert au nouvel exploitant, dans le même bassin d'emploi et dans le même métier. Une telle solution garantirait un seuil minimal d'acceptabilité sociale de l'ouverture anticipée à la concurrence. En favorisant la responsabilisation du salarié,